monsieur le président.

Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers qui doivent tenir compte du droit local, ce qui a des conséquences fiscales et sociales sur les relations entre ces établissements et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Pour ces raisons, le développement d'un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d'une entité juridique distincte. Cette entité est alors liée contractuellement ou statutairement à l'établissement scolaire. Malheureusement, dans ce type de situation, le dispositif proposé, comme celui auquel il se substitue, ne permet pas de demander une garantie de l'État, alors que celle-ci peut se révéler indispensable pour réaliser le projet immobilier dans des conditions financières raisonnables.

l'octroi de la garantie de l'État aux entités juridiques liées aux établissements français d'enseignement à l'étranger. Il ne me paraît pas que ce soit à l'État d'apporter sa garantie aux entités juridiques qui ne sont pas des établissements français d'enseignement à l'étranger.

puissent participer, aux côtés de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à l'instruction des demandes de garantie. Quel est l'avis de la commission mon cher collègue. Néanmoins, le nouveau dispositif proposé pour l'octroi des garanties prévoit que l'avis sur l'octroi de la garantie de l'État soit confié à une commission interministérielle, dont la composition sera précisée par décret.

réfléchissait déjà à la meilleure façon d'intégrer les parties prenantes, notamment les associations de parents d'élèves. Par ailleurs, votre demande me semble en partie satisfaite, puisque l'évaluation préalable du présent article indique que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger participera à l'instruction des dossiers. Je sollicite le retrait

totalement » -dérogatoire au droit commun, aux règles prudentielles et aux règles relatives au monopole bancaire. Les règles régissant ce nouveau dispositif doivent lui permettre d'être compatible la réglementation européenne en matière d'aides d'État, à laquelle personne ne peut se soustraire. Ces règles édictées par la Commission européenne sont très claires : pour ne pas être considérée comme une aide d'État, une garantie ne doit pas couvrir l'intégralité du prêt.

l'avis du Gouvernement

soit l'établissement situé à l'étranger empruntait auprès d'une banque et obtenait la garantie de l'Anefe pour le compte de l'État ; soit c'est cette dernière qui empruntait et qui consentait ensuite un financement à l'établissement scolaire au même taux que celui auquel il empruntait,

Il est certain qu'il est moins risqué pour une banque de consentir un financement à un lycée qui se trouve en Belgique plutôt qu'à un lycée qui se trouve en Guinée. Or l'objectif premier de ce dispositif est d'aider ceux des établissements qui ont le plus de difficultés pour emprunter sur le marché.

est à M. Bernard Buis. Cet amendement a pour objet de fixer à 0,5 % le taux maximum de la commission rémunérant la garantie de l'État aux projets immobiliers des établissements français d'enseignement à l'étranger. Le taux de la commission s'élève actuellement à 0,4 %. Il s'applique de manière uniforme à l'ensemble des établissements bénéficiant de la garantie de l'État par l'intermédiaire de l'Anefe.

Cette dernière doit donner lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché. Or le prix du marché doit inclure le risque encouru par l'État, et ce risque dépend effectivement du pays où se situe l'établissement français d'enseignement à l'étranger. Au reste, même hors cadre européen, il me paraît judicieux que la rémunération de l'État tienne compte du risque qu'il prend. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionnent tous nos dispositifs de garantie. J'émets

dans la foulée de l'accord de Paris, les dirigeants des pays du G20 se sont une nouvelle fois engagés à sortir des subventions aux énergies fossiles, mais les actes tardent. dans le présent article- 2025 pour le pétrole, 2035 pour le gaz -démontrent un manque d'ambition en contradiction avec les objectifs climatiques que s'est fixés la France. Nous ne pouvons que regretter la faible portée normative de ces trajectoires lointaines, alors que le Royaume-Uni prévoit d'annoncer prochainement l'arrêt net de ses crédits export aux énergies fossiles.

Pour empêcher un transfert de la production de ces pays vers le charbon, bien plus émetteur de gaz à effet de serre, et pour empêcher que les populations de ces pays n'en fassent les frais par une baisse du pouvoir d'achat, il est essentiel de réfléchir au plus vite aux moyens de mobiliser notre politique d'aide publique au développement pour compenser pour compenser l'arrêt de ces subventions. C'est une des conditions de notre volontarisme. C'est pourquoi nous demandons la remise d'un rapport concernant les différents leviers en matière d'aide sociale et d'aide à la transition énergétique que peut mobiliser la France en la matière pour accompagner concrètement un développement soutenable à l'international.

actes : on ne peut pas, en même temps, affirmer la volonté de laisser dans le sous-sol l'essentiel des énergies fossiles et prolonger, jusqu'en 2025 pour le pétrole et jusqu'en 2035 pour le gaz,

sans filtre la proposition d'une « réduction, puis suppression des garanties à l'export pour les projets liés aux énergies fossiles », telle qu'elle a été formulée par la Convention citoyenne. L'amendement On ne peut pas le nier : il est quand même perturbant de constater les deux visages de la politique française en matière d'écologie. D'un côté, la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures était, selon le Gouvernement, un signal fort, un engagement dans la continuité de l'accord de Paris ; la France, disait-il, assume son rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Bref, il s'agissait d'un florilège d'autosatisfaction et d'autofélicitations ! De l'autre, la France continue, respectivement jusqu'en 2025 et 2035, de couvrir les prêts octroyés en vue d'exporter des biens et services ayant

Vous me direz probablement que ces mesures anti-climat sont documentées par un rapport ; cela tombe bien. Ce rapport repose sur une méthodologie déplorable : un questionnaire distribué à 200 entreprises et seulement un quart de réponses obtenues ; un questionnaire relayé par les fédérations professionnelles et des questions complaisantes. Si vous demandez aux entreprises qui réalisent un important chiffre d'affaires à l'export si elles souhaitent que l'État garantisse une large part de leurs activités, elles répondront oui, évidemment ! Ce rapport a toutefois le mérite de mettre en lumière que l'État se substitue aux banques privées qui refusent de garantir les cautions de soumission ou de bonne exécution. Il y a une faille de marché pour ces activités polluantes, tout comme ces activités engendrent des failles sismiques et les séismes induits de la déforestation. Au total, quatre projets soutenus entre 2015 et 2019 représentent 97 % des 4,5 milliards d'euros d'engagements au d'assurance-crédit. Mes chers collègues, voici quels sont ces projets, au confluent de la politique économique et de la diplomatie, mais bien loin des enjeux environnementaux : la construction et la mise en service d'un gazoduc entre la frontière turco-grecque et la mer Adriatique ; le développement d'un champ sous-marin et d'une unité flottante de liquéfaction et de stockage de gaz naturel au large du Mozambique ; deux programmes de création d'installations de liquéfaction

En effet, l'arrêt du soutien public à l'export aux filières gazière et pétrolière aura indéniablement un impact sur l'activité et l'emploi en France, une moindre

Cozic. Vous le savez, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain appelle à un changement complet de paradigme en matière d'aides publiques. Il ne s'agit pas de freiner l'activité économique, mais de rappeler que, quand l'État s'engage financièrement, il est en droit de poser ses conditions. conditions. Cet amendement vise à subordonner les aides publiques aux entreprises de plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires aux engagements écologiques et sociaux suivants : publier un bilan carbone de l'entreprise respecter une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ne pas délocaliser d'emploi si cela entraîne une baisse de la masse salariale publier des indicateurs de performance sociale ; atteindre un objectif de réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes ; se doter d'un plan de vigilance. Le non-respect de ces engagements serait passible d'une amende d'un montant équivalent aux aides perçues par l'entreprise majoré de 2 % de son chiffre d'affaires. Les deux amendements

En contrepartie des aides versées en vertu du présent texte, les entreprises seraient tenues d'adopter et de publier dans les six mois suivant la réception de l'aide un « rapport climat » comportant trois documents un bilan carbone renforcé et standardisé ; une stratégie climat articulée autour d'une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l'année 2021 et à horizon de 2030 ; un plan d'investissement permettant de mettre en oeuvre cette stratégie en tenant compte des effets sur l'emploi. Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l'évolution des postes d'émission significatifs chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées. Outre une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d'investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l'environnement et être en cohérence avec l'objectif global : garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° Celsius. L'entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée. À ce titre, nous défendons un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l'argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. Si l'État a le devoir de protéger ses entreprises, il a aussi celui de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir

octroyées dans le cadre du plan de relance d'accorder des dividendes et des rachats d'actions à leurs actionnaires et des bonus à leurs mandataires sociaux durant l'année 2021. Le Gouvernement mobilise un plan de relance exceptionnel à destination des entreprises. Il serait incompréhensible qu'un seul euro d'argent public soit utilisé pour rémunérer les actionnaires et les dirigeants des entreprises. Ils doivent être mobilisés pour maintenir les activités essentielles, l'emploi et les investissements, en particulier dans la transition écologique.

Le dispositif proposé pourrait ainsi avoir pour conséquence de retarder le déploiement des mesures du plan de relance, au risque d'en diminuer l'efficacité. L'amendement prévoit bien que l'accord peut être mis en place en 2021, mais, alors, le bénéfice des aides

Malgré les engagements à l'autorégulation des industries agroalimentaires et l'interdiction de la publicité pendant les programmes jeunesse des chaînes publiques, l'ampleur du marketing alimentaire pour des PGSS en direction des enfants se maintient, en particulier à la télévision et sur internet. Aussi, l'OMS, l'OCDE et la Commission européenne recommandent la mise en place d'un encadrement et d'une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants. Cet amendement vise, dans cet esprit, à imposer une taxe sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes. Cette taxe serait progressive et fonction de l'éloignement des produits par rapport aux recommandations nutritionnelles ; elle serait endossée par l'industrie agroalimentaire qui produit ces aliments. Les fonds récoltés seraient entièrement consacrés à la promotion d'une alimentation saine et durable dans le cadre du programme national de l'alimentation et de la nutrition. Quel

Enfin, l'identification des dépenses de promotion peut-être difficile dans un certain nombre de contrats complexes. C'est pourquoi je renouvelle l'avis défavorable

Les formules de rémunération par attribution de titres d'entreprise, assorties d'incitations fiscales, se sont donc développées. Le présent article en fait partie : il étend aux entreprises de taille intermédiaire l'exemption dont disposent déjà les jeunes PME en cas de distribution d'actions à leurs salariés ce mécanisme semble se substituer à une véritable revalorisation salariale. Le problème, mes chers collègues, c'est que les coûteuses et piteuses politiques d'allégement de charges- selon le discours consacré -ont fait la démonstration de leur pertinence limitée il a suffi que l'on déclenche le confinement pour que 700 000 à 800 000 salariés en CDD, en intérim ou en contrat précaire perdent leur emploi, quasiment du jour au lendemain, venant grossir les rangs des chômeurs dépourvus de toute activité. Rien ne permet de penser que la situation sera redressée avant le second semestre de 2022, maintenant que le consensus des économistes se fait sur une croissance pour 2021 ne permettant pas de remonter la pente glissante sur laquelle notre économie s'est s'est trouvée cette année. La sécurité sociale n'a pas vocation à être la variable d'ajustement des politiques salariales des entreprises. Il convient donc de la financer avec les moyens nécessaires, issus du partage de la richesse produite par le travail. Tel est le sens de cet amendement. Quel est l'avis

renchérir le coût du dispositif et n'apparaît pas nécessaire compte tenu du régime fiscal et social déjà applicable aux versements de l'intéressement sur un plan d'épargne salariale.

n° II-39 rectifié. La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Le secteur viticole représente 500 000 emplois directs et indirects en France. Les viticulteurs estiment que la crise a engendré un manque à gagner supérieur à 1,5 milliard d'euros. Or, à l'inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n'ont pas eu recours, dans leur très grande majorité, au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour poursuivre l'entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir. Les marchés et les salons sont annulés, les restaurants fermés et les exportations sont au ralenti. Il faut ajouter à cela le conflit entre l'Europe et les USA sur l'aéronautique, dont la filière vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, qui représente leur premier marché à l'export. L'enchaînement de ces crises a des répercussions considérables sur l'ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées, sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants. Tout cela se traduit par une baisse de leur chiffre d'affaires sur l'année 2020. Cette situation pourrait rendre très difficile le paiement des salaires et des charges en 2021. Afin de soutenir l'emploi dans ces exploitations, cet amendement vise à accorder une aide aux employeurs qui ont subi une baisse d'au moins 20 % de leur chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale. Cette aide, dont le montant serait égal à 10 % de la masse salariale 2020, serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient bien évidemment

n° II-40 rectifié. Cet amendement vise à tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir certains agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d'opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l'année 2020. Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Ainsi, pour avoir un effet, l'option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l'année doit aussi pouvoir s'appliquer en 2021. À défaut, l'exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l'année 2020 reflète davantage l'activité de l'année 2019, et dont la baisse d'activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l'activité d'avant la crise, ce qui serait très difficile à supporter. Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains constitue le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques de la covid sur le secteur agricole.

cet article n'a pas vocation à refinancer des prêts bancaires existants, sinon cela se traduirait par un transfert du risque des banques vers l'État. Cet amendement vise à inscrire au niveau législatif la règle selon laquelle l'octroi des prêts et la souscription d'obligations se font sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue de développer l'activité, par parallélisme avec ce que prévoient les règles d'encadrement des aides d'État pour le financement des risques.

conformément à une demande de la Commission européenne. Pour autant, les négociations sont encore en cours quant aux paramètres du dispositif, et les amendements proposés préemptent largement leur résultat, ce qui ne

vise à instaurer un plafond de financement par entreprise correspondant au plus petit montant entre le plafond en pourcentage du chiffre d'affaires prévu pour la dette

soixante-quatorze ans. Cette situation est profondément inéquitable pour les quelques-unes qui, hélas, ont vu leur conjoint décéder avant de pouvoir bénéficier de sa retraite.

est à M. Stéphane Artano. La viticulture française souffre gravement des conséquences de la crise sanitaire, à laquelle s'ajoute la surtaxation de 25 % imposée par les États-Unis sur les importations de vins français dans le cadre du conflit commercial opposant Airbus et Boeing. D'après les estimations du secteur, cette mesure tarifaire a déjà causé environ 400 millions d'euros de pertes : une gageure pour les professionnels et une vraie menace pour la vitalité de nos territoires viticoles.

vin et eau-de-vie de vin pour demander la mise en place d'un tel fonds. Pourtant, à ce jour, rien n'a été fait pour soutenir ces entreprises. Nous connaissons tous le goût

des régimes spéciaux à raison d'un congé maladie directement lié au covid. Nous voterons ce dispositif équitable et de nature à mieux protéger les agents publics dans la période en

mais se heurtent à des difficultés liées aux caractéristiques de leur territoire : des formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, un centre urbain extrêmement dense, un habitat vertical fortement présent. Cet amendement vise à leur donner la possibilité de mettre en place

il eût peut-être été préférable, pour faire gagner du temps à tout le monde et du calme dans les intercommunalités, de ne pas faire tout et n'importe quoi au moment des fusions d'intercommunalités, avec des remontées de compétences à marche forcée ... Texte après texte,

Le PLFR 3 a élargi le champ des entreprises éligibles à la réassurance de la Caisse centrale de réassurance aux grandes entreprises et aux risques d'assurance-crédit à l'export. Aujourd'hui, seules les entités françaises d'une entreprise française peuvent bénéficier de ces mesures. Or les emplois situés en France dépendent souvent également des ventes réalisées par les filiales étrangères de ces entreprises françaises. Cet amendement vise à permettre aux filiales de ces sociétés établies en France de bénéficier du dispositif de soutien public d'assurance-crédit à l'export CAP France export. Quel

ou leurs filiales étrangères situées en France et qui participent à l'économie nationale. Vous souhaitez l'étendre aux entreprises ayant souscrit leur

monsieur le ministre.

? Favorable. Je consulte le Sénat sur la demande de coordination, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission. Il n'y a pas d'opposition ? conformément à l'article 43, alinéa 5, du règlement, lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

362, « Écologie » et 363, « Compétitivité », en revenant sur la création du programme « Plan pour l'égalité réelle en outre-mer

550 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour l'action n° 05, Culture, du programme 363, « Compétitivité

taxe exceptionnelle sur les hauts revenus, taxe sur les géants du numérique, barème progressif de l'impôt sur les sociétés ... Je vous rassure, mes chers collègues, je ne vous réciterai pas la liste des amendements que nous avons déposés sur cette

sur une analyse de la réalité sociale dans notre pays. Nous nous abstiendrons sur cet amendement, car, ce qu'il prend aux Ultramarins, il le rend à l'écologie.

la procédure nous oblige à délibérer sur cet article d'équilibre, en attendant que la navette nous permette d'aboutir, quelle que soit l'appréciation que chacun portera sur le budget définitivement adopté, à un État qui puisse bénéficier des crédits pour l'ensemble des missions. Quel est l'avis de la commission